ce matin, au cours d'une conférence de presse, la préfecture de Seine-Maritime a voulu rassurer la population en indiquant que, malgré une odeur déplaisante d'hydrocarbures, la fumée et les suies ne présentaient « pas de toxicité aiguë Pourtant- c'est le fameux « en même temps » -, le préfet a également précisé que les écoles resteraient fermées par précaution, le temps de nettoyer les traces de suie. Ces éléments semblent profondément contradictoires, et l'inquiétude relative aux suites de l'incendie demeure au sein de la population. Madame la secrétaire d'État, la gestion par les pouvoirs publics d'un tel événement doit faire l'objet d'une transparence exemplaire, et la population doit être parfaitement informée des risques pour elle-même et pour l'environnement, notamment

un retour aux sols de haute qualité de différents flux de déchets organiques au travers du compostage. Ce compostage doit s'effectuer en toute sécurité et répondre aux exigences suivantes : ne concerner que des déchets non dangereux contenant principalement de la matière organique et pouvant, à l'état brut, faire l'objet d'une valorisation agronomique ; faciliter leur réemploi et conduire à la production de matières fertilisantes dont les critères de qualité et d'innocuité sont conformes à un règlement européen, une autorisation de mise sur le marché, à une norme rendue d'application obligatoire ou à un cahier des charges, la traçabilité devant être assurée à toutes les étapes du traitement et, le cas échéant, jusqu'aux parcelles d'épandage. Il s'agit donc de promouvoir et de sécuriser la filière de retour aux sols des matières organiques issues de l'économie circulaire, en offrant aux utilisateurs et aux citoyens toutes les garanties nécessaires en termes de sécurité sanitaire et de protection de l'environnement.

l'amendement n° 231 rectifié . Les évolutions de la réglementation relative à la valorisation des matières fermentescibles inquiètent beaucoup d'acteurs du secteur et remettent en cause nombre de projets de valorisation par méthanisation ou compostage. L'un des enjeux est notamment la possibilité de mélanger certains flux de matières fermentescibles dans des opérations de valorisation. En effet, le Gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent ainsi pas être mélangés avec d'autres matières fermentescibles. Les mélanges de matières fermentescibles issues du traitement des eaux- boues d'épuration, notamment -avec d'autres flux sont également remis en question. Il est important de garantir au maximum la qualité et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Toutefois, la logique appliquée jusqu'ici exclut aveuglément certaines matières en fonction de leur origine, et empêche le développement de plusieurs types de projets de valorisation organique qui pourraient pourtant produire des matières fermentescibles respectant les normes de qualité et d'innocuité appliquées aux intrants agricoles. Le compostage des boues d'épuration nécessite également un apport de structurants sous forme de déchets verts, afin d'améliorer les conditions de biodégradabilité des boues : porosité, équilibre de l'humidité, apport de carbone. Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent les filières de ce type. Les déchets concernés risquent donc de quitter l'économie circulaire pour entrer dans l'économie linéaire,

Cet amendement vise donc à préciser l'amendement adopté par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable prévoyant un décret définissant les conditions dans lesquelles les boues peuvent être traitées conjointement avec d'autres matières par compostage. Il tend à préciser que ce procédé doit pouvoir permettre la production d'un compost

Ces nouvelles réglementations écartent par ailleurs certaines matières fermentescibles, uniquement en fonction de leur origine. Cet amendement vise donc à prévoir l'élaboration d'un décret définissant les conditions dans lesquelles les boues peuvent être traitées conjointement avec d'autres matières. Il tend à préciser que ce procédé doit rendre possible la production d'un compost conforme aux normes de qualité permettant son retour aux sols. Afin de garantir au maximum la sécurité des sols, cette mesure pourrait être accompagnée d'un renforcement de normes permettant le retour aux sols des matières fermentescibles

et ne permet pas de garantir que ces matières soient bien organiques. Cela signifie par exemple que les cartons, qui contiennent des substances toxiques, notamment dans les encres, pourraient entrer dans la composition des composts. L'objet de cet amendement est de permettre le maintien de la filière de compostage conjoint des boues de stations d'épuration et des déchets verts, tout en s'assurant de la qualité des matières entrantes. Si le mélange de déchets présente un intérêt pour les opérations de collecte et de traitement, il soulève de nombreux problèmes pour la valorisation en agriculture : un risque inacceptable de pollution des sols et d'insécurité sanitaire des aliments du fait de la qualité inconnue des matières entrantes une surface agricole polluée plus importante en cas de problème post-épandage ; une perte de traçabilité du fait des origines diverses des déchets, complexifiant la définition de la responsabilité en cas de problème post-épandage. L'évolution vers une économie circulaire ne doit pas être au détriment de la sécurité sanitaire des aliments et de la gestion des risques environnementaux.

des déchets a, entre autres objectifs, celui d'« augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse [ ...] pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés ». En lien avec la mise en place de ce dispositif fort, le Gouvernement a introduit dans la réglementation des interdictions de mélange de certains flux de déchets. Ainsi, les biodéchets des ménages collectés séparément ne peuvent pas être mélangés avec d'autres matières fermentescibles. Évidemment, il est important de garantir la qualité et l'innocuité des matières fermentescibles utilisées sur nos sols, et de ne pas gâcher le geste de tri des Français dont les biodéchets ont été collectés séparément. Cependant, la logique appliquée ici frontalement exclut certaines matières en fonction de leur origine et empêche le développement de projets de valorisation organique visant à produire des matières fermentescibles qui respectent les normes de qualité et d'innocuité propres aux intrants agricoles. Par exemple, le compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles nécessite l'apport de structurants- le plus souvent sous la forme de déchets verts -pour assurer les conditions de biodégradabilité. Les restrictions réglementaires sur les mélanges de biodéchets excluent donc les filières de ce type. Les déchets concernés risquent ainsi de quitter l'économie circulaire pour entrer dans une économie linéaire. Cette situation est en totale contradiction avec les objectifs de la France en matière d'économie circulaire et de réduction du stockage des déchets. C'est pourquoi nous présentons cet amendement, qui vise à préciser que les déchets verts peuvent être utilisés comme structurants dans le processus de compostage de la fraction fermentescible issue du tri des ordures ménagères résiduelles, à condition que le compost produit ainsi respecte les normes d'innocuité en vigueur. Sont exclus tous mélanges de biodéchets ménagers issus de la collecte séparée, afin de ne pas gâcher le geste de tri des ménages. La parole est à Mme Christine Lavarde,

de la commission ? La commission a introduit une base législative permettant d'assurer le maintien du compostage en mélange des boues d'épuration avec d'autres produits structurants dans des conditions fixées par voie réglementaire. La solution retenue en commission nous semblant plus équilibrée, je vous demanderai de bien vouloir retirer vos amendements, mes chers collègues.

entre la classification des substances radioactives par les exploitants, d'une part, et les décisions prises par ces mêmes exploitants relatives aux charges et provisions de gestion de ces substances, d'autre part Cet enjeu concerne l'uranium dit « de retraitement » ainsi que les MOX usés. Ces derniers sont aujourd'hui considérés comme des « matières », car une valorisation est théoriquement envisagée.

réelles perspectives de valorisation, ces combustibles MOX sont comptablement traités par EDF comme des déchets et donnent lieu à un provisionnement et à une couverture par des actifs dédiés pour leur stockage, à hauteur de 656 millions d'euros.

Cet amendement vise à exiger une requalification des matières radioactives en déchets ultimes, au regard de leurs perspectives actualisées de valorisation. Il s'agit de choix profondément structurants pour la filière nucléaire. Nous partageons les inquiétudes de notre collègue sur le risque d'une éventuelle surévaluation des capacités de valorisation de certaines matières, d'une sous-évaluation des responsabilités en termes de fin de vie

pour l'évaluation des perspectives de valorisation des matières nucléaires et, le cas échéant, leur requalification en déchets. Il prévoit en effet qu'à chaque révision du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, les propriétaires de matières radioactives informent les ministres chargés de l'énergie et de la sûreté nucléaire des procédés de valorisation qu'ils envisagent. C'est sur la base de ces informations que les ministres peuvent être amenés à prendre une décision de requalification. Toutes les matières disposent aujourd'hui de perspectives de valorisation. S'agissant, par exemple, des combustibles MOX usés, le Gouvernement a réaffirmé, dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, son engagement à poursuivre une stratégie du cycle fermé il a fixé un objectif intermédiaire de multirecyclage des combustibles MOX usés en réacteur à eau pressurisée à l'horizon 2040. Un programme de recherche et développement dédié à cet objectif doit être mis en oeuvre par la filière. Le Gouvernement a bien pris note de la recommandation de la Cour des comptes relative à la transparence du processus de décision conduisant à requalifier une matière en déchet et a souhaité soumettre cette question au débat public en cours sur les matières et déchets radioactifs en ouvrant plusieurs pistes

de réacteurs, dont le Gouvernement a annoncé officiellement l'abandon cet été. Des perspectives théoriques pourraient se dessiner à long terme,

Cet amendement vise à favoriser l'exploitation et le développement d'installations vertueuses de traitement des déchets en privilégiant les déchets non valorisables issus des filières de recyclage par rapport aux déchets non triés en amont.

la filière CSR pourrait consommer efficacement certains déchets ultimes aujourd'hui envoyés à l'enfouissement. La valorisation énergétique des combustibles solides de récupération permettant de produire de la chaleur ou de l'électricité en substitution de ressources fossiles, elle représente une solution particulièrement intéressante. La France doit donc donner une impulsion politique forte à la consommation de combustibles solides de récupération et exploiter le potentiel

Il est urgent de mettre en place des mesures fortes, garantissant l'acceptation des déchets non valorisables dans les conditions techniques et économiques du moment.

des déchets au niveau des opérateurs économiques. En effet, actuellement, l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement, issu de la loi pour la transition énergétique de 2015, prévoit la définition des modalités d'application du tri obligatoire cinq flux dans les entreprises, mais pas les modalités de suivi et de contrôle.

est à Mme Laure Darcos. La lutte contre les dépôts sauvages de déchets est devenue une priorité des élus locaux, de plus en plus confrontés à ce type d'incivilités qui non seulement portent atteinte à l'environnement, mais aussi pèsent lourdement sur les budgets des collectivités locales.

Le présent amendement vise à instaurer, en cas de récidive, une peine complémentaire de confiscation du véhicule ayant servi à transporter les déchets, matériaux et autres objets abandonnés, jetés ou déversés illégalement.

Aujourd'hui, aucune expérience dans le monde ne permet de penser que le stockage souterrain est absolument sûr, fiable et durable à long terme. La Belgique

Cet amendement vise à définir la notion de reconditionnement, afin de créer de la confiance sur un marché en plein, mais dont l'essor pourrait être freiné par le manque de confiance des clients. En effet, à ce jour, aucun texte législatif ou réglementaire n'encadre cette notion,

D'autres ont fait l'objet d'une analyse méticuleuse de chaque pièce, mais sans remplacement systématique. Cette confusion nuit au marché du reconditionnement, qui nécessite de la confiance.

vise à faire émerger une mention signalant les produits qui bénéficient de la meilleure qualité de reconditionnement, afin de les valoriser. Il s'agit de rassurer le consommateur lors de son acte d'achat, en lui certifiant que le produit reconditionné respecte certains critères de qualité qui seront définis par décret.

Les reportages dénonçant l'exportation de déchets produits en France se multiplient. Les citoyens sont alertés sur cette question et ils la prennent à coeur, estimant à juste titre que les pays d'Asie et d'Afrique ne doivent pas avoir à gérer les déchets produits par les pays riches. Il faut les écouter et agir en conséquence. La décision de la Chine de mettre fin au début de 2018 aux importations de déchets a suscité le chaos sur le marché mondial du recyclage et a obligé les pays développés à trouver de nouvelles destinations pour leurs déchets. En 2018, c'est entre 450 000 et 700 000 tonnes de déchets qui ont été exportées chaque mois vers la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines et d'autres pays d'Asie. On ne fait que déplacer les problèmes dans des pays où les plastiques et déchets en tout genre sont « recyclés » de manière très artisanale, c'est-à-dire le plus souvent brûlés sans aucune précaution pour l'environnement et la santé des habitantes et des habitants. Ils finissent aussi souvent par polluer les eaux. Depuis le mois de juin 2019, l'Indonésie a d'ailleurs renvoyé plusieurs centaines de conteneurs de déchets non conformes vers leur pays d'origine. Sur l'île indonésienne de Batam, proche de Singapour, quarante-neuf conteneurs de déchets non conformes ont ainsi été saisis et renvoyés vers les États-Unis, l'Allemagne, Hong Kong et la France.

Alors que le projet de loi initial renvoyait ce sujet très important à des ordonnances, la commission a considéré qu'il appartenait au législateur d'en débattre et de décider des meilleurs outils pour lutter contre ce fléau. Elle a donc introduit plusieurs dispositions visant à lutter en amont contre ces dépôts sauvages. En premier lieu, les mesures prévues pour la gestion des déchets du bâtiment permettront de lutter contre les dépôts sauvages de déchets, largement constituées de déchets issus Par ailleurs, des dispositions dont nous avons déjà discuté permettront que les éco-contributions versées par les producteurs contribuent à financer le nettoyage des dépôts sauvages. En plus de ces mesures préventives et curatives, la commission a souhaité intégrer plusieurs dispositions répressives dans un nouveau titre consacré à la lutte contre les dépôts sauvages. Elle a prévu de donner la faculté aux maires de transférer au président de leur EPCI leurs pouvoirs en matière de lutte contre ces dépôts. Nous avons également entendu habiliter les agents de surveillance de la voie publique et des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions déterminées par voie réglementaire à constater les infractions relatives aux dépôts sauvages. également instauré des sanctions en cas de non-respect du tri cinq flux par les entreprises. En outre, la commission a donné accès au système d'immatriculation des véhicules aux personnes habilitées à rechercher et à constater les infractions liées à l'abandon ou au dépôt illégal de déchets. Elle a permis la vidéoverbalisation des auteurs de dépôts sauvages. La commission a également prévu d'obliger les derniers usagers d'un véhicule à produire un certificat de destruction d'un véhicule hors d'usage lors de la déclaration de cessation de l'assurance.

ces précisions très importantes. Madame la secrétaire d'État, lors de votre audition par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, je vous avais fait part du sentiment d'impuissance des maires ruraux face aux dépôts sauvages de déchets, dont ils sont dans l'impossibilité de sanctionner les auteurs. auteurs. Si de telles infractions peuvent être sanctionnées sur le plan pénal, les plaintes sont, dans la grande majorité des cas, classées sans suite par le procureur.

distinguer la procédure pour les atteintes majeures à l'environnement, relevant des services de l'État, et la lutte contre les dépôts sauvages, relevant de la compétence des maires. Dans le second cas, afin que l'intervention puisse être rapide,

L'attente est forte dans nos territoires, et ces amendements identiques visent à y répondre le plus rapidement possible. L'avis de la commission est donc favorable.

Je ne voudrais pas être désagréable, mais tout de même : j'ignore si les amendements sont satisfaits, mais je sais que, avec les dispositions actuelles, les maires, eux, ne sont pas satisfaits

qu'elles ne font pas qu'enlever les déchets des ménages ; elles enlèvent également les déchets assimilés, comme les déchets sauvages et les encombrants. Cette question n'est pas uniquement juridique, mais aussi financière, parce que la possibilité d'affecter le

L'article L. 2224-14 du même code prévoit que les collectivités territoriales assurent la collecte des déchets assimilés, définis comme les déchets d'activités économiques qu'elles peuvent prendre en charge dans les mêmes conditions que les déchets des particuliers. L'objectif est d'étendre le périmètre du service public aux déchets qu'il est difficile de différencier des déchets ménagers, tout en éliminant cette extension pour prendre en compte la dimension concurrentielle avec le secteur privé pour la gestion des déchets. Pour moi, cette définition des déchets assimilés

les dépôts sauvages. Il a mis en lumière la détresse des élus face à des situations difficiles. Les pouvoirs de police du maire doivent être renforcés. Aujourd'hui, l'article L. 541-3 du code de l'environnement définit la procédure de sanction

Selon un rapport de l'Ademe, en l'absence de mécanismes financiers de compensation, les coûts pèsent majoritairement sur les collectivités territoriales. Cette étude a révélé, sur la base d'un questionnaire, qu'ils s'élèvent en moyenne à plus de 59 000 euros

d'encourager les professionnels du BTP à utiliser ces équipements. Mon propos n'est pas de stigmatiser, mais d'accompagner les artisans, qui se retrouvent souvent sans réelle solution pour déposer les gravats. Si nous pouvons nous féliciter du maillage de nos décharges

maires détiennent en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, s'agissant de la collecte des déchets ménagers, aux présidents de groupe de collectivités territoriales au sens large, et non uniquement aux présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre,

En tout état de cause, afin de lutter efficacement contre les dépôts sauvages de déchets ménagers, toutes les possibilités doivent être ouvertes pour permettre aux élus et aux autres acteurs locaux de répondre

sur le fondement de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, lorsque le véhicule peut être considéré comme un déchet ; dans le cas où le véhicule n'est pas retiré dans le délai imparti, le maire peut faire procéder d'office, aux frais de son propriétaire, à l'exécution des mesures prescrites.

d'éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation ou lorsque sa circulation ou son stationnement contrevient à la sécurité, à l'esthétique ou au passage, il n'est pas précisé si les frais d'enlèvement peuvent être mis à la charge du propriétaire du véhicule hors d'usage. Or les frais de mise en fourrière, de retrait de la circulation ou de destruction peuvent être importants pour les communes. Cet amendement a donc pour objet de préciser

sont cependant à la charge de l'autorité dont relève la fourrière, c'est-à-dire l'État ou les collectivités territoriales, lorsque le propriétaire du véhicule s'avère inconnu, introuvable ou insolvable.

Mme Jacky Deromedi. Depuis plusieurs années, nous assistons à la multiplication des systèmes de vidéosurveillance dans les communes françaises. Ceux-ci ont montré leur efficacité en bien des endroits et dans de nombreuses affaires. Les Français sont nombreux à ressentir une véritable exaspération à la vue de déchets abandonnés en pleine nature, gâchant la pureté d'un paysage et polluant les lieux dans un contexte où le traitement des déchets est une priorité face au réchauffement climatique et à l'avenir incertain de notre planète. Le drame du maire de Signes, décédé dans l'exercice de ses fonctions en tentant d'interpeller deux individus en train de déposer illégalement des ordures, est insupportable pour les élus Si la loi du 24 juillet 2019 a amené une grande avancée en matière de lutte contre ces dépôts illégaux, en permettant la transmission d'images de vidéosurveillance aux autorités publiques en vue de signaler l'abandon d'ordures, rien à ce jour ne permet la permet la verbalisation à distance par ce type de système. Pourtant, les dépôts illégaux de déchets sont, pour la plupart, effectués au moyen d'un véhicule.

qui a pour objet de lutter contre les filières illégales de traitement de véhicules hors d'usage. De fait, 500 000 véhicules seraient traités et, parfois, exportés illégalement chaque année, en raison de la valeur résiduelle positive de leurs pièces détachées et de leurs métaux. Ce sont ainsi des centaines de milliers de tonnes de matières recyclables- métalliques ou plastiques -qui ne sont pas mises à disposition des filières françaises de recyclage. Les conditions de traitement des véhicules dans les sites illégaux peuvent par ailleurs conduire à des pollutions de l'environnement- absence de récupération des huiles, des liquides de toute nature, des gaz de climatisation, etc. Le présent amendement vise à consolider l'efficacité du dispositif dans le cas de véhicules endommagés considérés comme techniquement ou économiquement irréparables par la société d'assurance. Il tend à imposer que le propriétaire d'un véhicule non réparable qui refuse la reprise et l'indemnisation par la société d'assurance fournisse à ladite société un justificatif de destruction dans une installation dûment autorisée. En l'absence de justification, le propriétaire continuera de payer sa cotisation tant que le certificat de destruction ne sera pas remis, ce qui l'incitera à faire procéder à la destruction dans une installation légale.

L'alinéa 3 de l'article 12 G impose aux professionnels chargés des travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments de transmettre au maître d'ouvrage un certificat qui atteste que les déchets ont été collectés ou traités conformément aux informations inscrites dans le devis. Une telle obligation est, dans les faits, compliquée à satisfaire. En effet, les artisans ne déposent pas systématiquement les déchets produits à l'issue de chaque chantier. Pour des raisons évidentes de logistique, l'entreprise doit limiter ses déplacements et elle regroupe les déchets issus de plusieurs chantiers. Si les entreprises doivent être en mesure de justifier de la traçabilité des déchets, l'obligation d'établir un certificat à la fin du chantier semble peu appropriée à la pratique. Le présent amendement a pour objet de prévoir l'obligation pour les entreprises de justifier de la traçabilité des déchets.

Afin de lutter contre les dépôts sauvages de déchets, l'obligation pour les professionnels du bâtiment de présenter à leurs clients un certificat attestant de la prise en charge des déchets a été introduite en commission. Toutefois, ce dispositif n'est assorti d'aucune mesure d'obligation ni même d'incitation, et il n'est pas prévu, dans la rédaction actuelle, que son non-respect entraîne des sanctions. Cet amendement vise donc à rendre la mesure plus efficace, en conditionnant

ils visent à supprimer l'obligation de remise au maître d'ouvrage d'un certificat de traitement des déchets, mesure que la commission avait unanimement soutenue. Or l'objectif est bien d'associer les maîtres d'ouvrage à la gestion des déchets afin qu'ils puissent s'assurer que ceux-ci ont été traités régulièrement et qu'ils n'iront pas alimenter les dépôts sauvages. La rédaction proposée par les auteurs de ces amendements limiterait l'efficacité de ce dispositif en matière de lutte contre les dépôts sauvages de déchets issus du secteur du bâtiment. Deuxièmement, le regroupement des déchets de plusieurs chantiers par les professionnels du bâtiment ne me semble pas faire obstacle à la mise en place de ce certificat, comme le soutiennent les auteurs de ces amendements.

Afin d'assurer une cohérence dans les actions engagées par les collectivités au regard tant de la propreté que du service public de gestion des déchets, le présent amendement tend à ouvrir la possibilité, pour les collectivités le désirant, d'intégrer la dimension de la propreté au service public

d'enlèvement des ordures ménagères. Lier la compétence de propreté à celle de traitement des déchets permet de relégitimer la participation des opérateurs privés aux missions de service public. La parole est à M. Claude

Un tel élargissement permettrait aux collectivités compétentes de prendre en compte le coût lié à la collecte et au traitement des déchets de rue dans la détermination du taux de leur TEOM. Une telle extension peut être Une telle extension peut être utile pour permettre aux collectivités de mieux financer leurs services de propreté et de collecte des déchets de rue. Mais, en augmentant la part fixe de la TEOM, elle pourrait avoir pour effet d'affaiblir les effets positifs de sa part incitative lorsque celle-ci a été mise en place. Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat sur les amendements identiques n

les arguments très convaincants avancés par Mme la rapporteure, j'indique que le service public de gestion des déchets n'intègre pas, à ce jour, le nettoyage des déchets abandonnés dans la rue,

Merci,

L'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales dispose que les collectivités locales assurent la collecte et le traitement des déchets d'activités économiques qu'elles peuvent « collecter et traiter sans sujétions techniques particulières La notion de sujétions techniques particulières est assez clairement définie par la jurisprudence : les déchets assimilés doivent pouvoir être collectés et traités en même temps et dans les mêmes conditions que les déchets ménagers, et donc par les mêmes installations. votre proposition ouvrirait totalement le périmètre du service public de gestion des déchets. Les collectivités pourraient traiter tout type de déchets pourvu qu'elles se dotent des installations nécessaires, y compris en entrant en concurrence avec une offre privée déjà existante. Je ne suis pas certaine que les collectivités territoriales disposent des moyens- en particulier des moyens humains

Une telle situation entraîne des incertitudes pour les professionnels qui utilisent le service public, en raison de grandes disparités constatées dans l'appréciation locale, par les collectivités territoriales, du caractère assimilé des déchets non ménagers, ainsi que des différentes composantes définissant le service public. Une définition incorrecte des déchets assimilés peut placer les collectivités locales en situation de risque juridique

? Actuellement, ce sont les collectivités territoriales elles-mêmes qui déterminent, dans leur règlement de collecte, quels déchets d'activités économiques elles peuvent collecter dans le cadre du service public de gestion des déchets. Cette situation est source de variété juridique, puisque les déchets collectés peuvent différer d'une commune à une autre et que les collectivités peuvent se retrouver en concurrence avec les opérateurs privés pour la gestion de ces déchets. Cependant, la fixation de seuils maximums que vous proposez est inappropriée : la situation particulière de chaque collectivité doit être prise en compte. Par exemple, l'organisation d'une métropole de plusieurs centaines de milliers d'habitants

En effet, la loi pour la transition énergétique de 2015 a modifié l'article L. 541-1 du code de l'environnement, en précisant que la généralisation du tri à la source des biodéchets en orientant ces déchets vers des filières de valorisation en matière de qualité rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, lequel doit donc être évité et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. Or de telles dispositions ne permettent pas de clarifier le devenir des installations concernées ainsi que les investissements devant être apportés par les différents acteurs. Compte tenu de ce manque de clarté, la loi a été interprétée de manière variée par diverses cours de justice. Aussi cet amendement a-t-il vocation à clarifier la disposition précitée, afin d'unifier la situation sur le territoire.

ni par la directive elle-même ni par la jurisprudence. La gestion des explosifs déclassés du ministère des armées est donc soumise à de lourdes contraintes administratives pour permettre le franchissement des frontières- notification et consentement préalable des États concernés -, ce qui n'est pas le cas dans les pays voisins. de traitement des déchets de ce type étant insuffisantes sur le territoire national, l'état actuel de la réglementation complexifie inutilement les missions du service interarmées des munitions du ministère des armées, sans aucun bénéfice pour la protection de l'environnement.

n° 93 rectifié. Cet amendement, issu d'une discussion avec l'Union nationale des exploitants du déchet, vise à introduire directement dans la loi un véritable statut des terres excavées afin de garantir un haut niveau de traçabilité permettant de prévenir les atteintes potentielles à l'environnement et à la santé humaine. Il est proposé de créer un statut particulier, intermédiaire entre le régime de droit commun des déchets et la sortie pure et simple du statut de déchet. Ce statut particulier, parfaitement compatible avec la directive-cadre européenne sur les déchets du 19 novembre 2008, pourrait être structuré autour des principes suivants. rendre obligatoire la réalisation d'un contrôle préalable de la qualité des terres par les personnes à l'origine de la décision d'excavation des terres- entrepreneurs, promoteurs, maîtres d'ouvrage, etc. Ce contrôle serait effectué sous la responsabilité du producteur des terres et par l'exploitant d'une installation classée- IOTA -, un expert agréé ou un organisme public indépendant. Ce contrôle donnerait lieu à la réalisation d'un rapport de qualité des terres qui contiendrait les informations permettant d'identifier le site d'origine, l'identité du maître d'ouvrage et du propriétaire, de connaître le volume et les caractéristiques des terres et de lister les usages théoriques possibles en fonction de la caractérisation préalable. En deuxième lieu, rappeler l'obligation d'un traitement préalable en installation classée autorisée des terres excavées impactées présentant des concentrations supérieures à des seuils qui devront être fixés par décret. Ce principe permet d'assurer la conformité à la directive-cadre sur les déchets, qui requiert que le traitement de déchets soit réalisé dans une installation soumise à autorisation ou,, à enregistrement. prévoir la réutilisation des terres excavées inertes ou devenues inertes après traitement, soit sur un site receveur soumis à ICPE ou à IOTA, pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction, soit sur tout type de site receveur pour des projets de construction, de génie civil ou d'aménagement certifiés. Enfin, encadrer la réutilisation des terres par le site receveur. Pour pouvoir être réutilisées sur un un site receveur, les terres devront respecter les seuils précités. Le propriétaire ou l'exploitant du site receveur devra non seulement réaliser une étude préalable permettant de garantir l'aptitude du site receveur à recevoir les terres excavées, mais également consigner le volume des terres excavées réutilisées pour en garantir la traçabilité. De manière dérogatoire, toute personne réutilisant des terres excavées respectant les seuils à des fins de réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction pourra recevoir une contrepartie financière pour l'utilisation de ces terres.

Cet amendement de repli a pour objet de faciliter la sortie du statut de déchet afin de permettre une meilleure réutilisation des déchets comme matières premières, dans une logique d'économie circulaire. Son adoption permettrait de favoriser les entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire spécialisées dans la réutilisation ou le réemploi des déchets. Cette facilitation de la sortie du statut de déchet doit toutefois être encadrée, afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine, conformément à la directive 2008/98 sur les déchets. Cet encadrement est nécessaire s'agissant en particulier des déchets dangereux qui peuvent présenter des risques pour la santé humaine ou l'environnement, ainsi que des terres excavées, dont une mauvaise gestion peut entraîner une migration de la pollution, une contamination ou une détérioration de la qualité des sols ou des eaux souterraines. C'est la raison pour laquelle

et à faciliter la sortie du statut de déchet non dangereux, qui peut désormais intervenir en dehors des installations classées, IOTA ou ICPE. Le fait, d'une part, de limiter le passage préalable en ICPE ou en IOTA aux seuls déchets dangereux et terres excavées, et, d'autre part, de faciliter la sortie du statut de déchet pour les déchets non dangereux est pleinement conforme à la directive, aux termes de laquelle les États membres doivent faciliter une « utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles

Le droit communautaire a instauré une procédure de sortie du statut de déchet pour faciliter la valorisation des déchets dans des conditions encadrées, permettant d'assurer la protection de l'environnement. La sortie du statut de déchet est donc un outil efficace de développement de l'économie circulaire. Aujourd'hui, la loi prévoit qu'elle ne peut avoir lieu que dans une installation relevant du régime des installations classées pour la protection de l'environnement. Or l'instauration de cette obligation est une surtransposition de la directive européenne Déchets. identiques permet de simplifier la procédure de sortie du statut de déchet tout en maintenant une procédure stricte pour les déchets dangereux. Je propose d'aller plus loin dans la simplification, tout en ajoutant la possibilité de faire appel à un tiers pour contrôler la procédure de sortie du statut de déchet, ce qui renforcera les exigences et la traçabilité de cette procédure. En effet, certaines installations présentent suffisamment peu d'enjeux pour ne pas être classées, comme une petite entreprise de l'économie sociale et solidaire qui répare des téléphones portables ou des réfrigérateurs. Dans ce cas, il est pertinent de lui permettre de récupérer et de vendre les objets réparés comme des produits. les terres excavées et sédiments pollués nécessitent un contrôle très rigoureux, exercé soit au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement, soit par des organismes tiers accrédités. Ces contrôles permettront également de renforcer la traçabilité du devenir des terres excavées. Nous travaillons notamment avec des ONG comme Robin des Bois pour garantir la rigueur de telles procédures.

non dangereux seulement, ce qui veut dire que les terres excavées présentant les caractéristiques de déchets dangereux ne pourront sortir du statut de déchet sans avoir été traitées dans une installation classée.

parole est à Mme Laure Darcos. Le présent amendement vise à préciser et à encadrer les dérogations ponctuelles, pour les arrêtés préfectoraux d'autorisation d'installations de traitement de déchets-principalement des installations d'incinération ou de stockage de déchets non dangereux-, aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets pris en application des dispositions de l'article L. 541-13 du code de l'environnement ou, dans les régions concernées, aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif continuera à permettre une gestion des déchets offrant le meilleur résultat sur le plan de l'environnement dans des situations locales dégradées, en particulier en cas de déficit de capacités locales de traitement, tout en garantissant que cette dérogation ne sera utilisée

Parmi ces derniers, la création d'une nouvelle installation de stockage de déchets non dangereux, non seulement prioritaire, mais aussi excessivement contrainte. Du fait de sa géographie et de son organisation administrative, la Guyane est particulièrement concernée par les dispositions de la loi Littoral. Sur les vingt-deux communes guyanaises, quatorze relèvent des dispositions de cette loi, alors même qu'elles concentrent la quasi-totalité de la population guyanaise et, partant, les besoins en équipements. Dans ce contexte, lorsque les contraintes liées au risque aviaire et à la loi Littoral se conjuguent pour ces communes, il ne reste plus aucune zone accessible susceptible d'accueillir une unité de stockage de déchets. défaut de dérogation à la loi Littoral sur l'obligation d'étendre l'urbanisation en continuité du bâti, la Guyane sera confrontée à une crise majeure à court terme. Le présent amendement a donc pour objet de prévoir une nouvelle dérogation à la loi Littoral. Chers collègues, je sais que le sujet est sensible. J'aimerais donc insister sur le fait que cet amendement est le fruit d'un travail de concertation de plusieurs mois, pour ne pas dire de plusieurs années, au niveau local. Nous sommes Nous sommes aujourd'hui au bout d'un processus, et toutes les parties prenantes, élus comme services de l'État, conviennent qu'une telle dérogation est devenue indispensable. J'ajoute que cette dérogation apparaît d'autant plus opportune que la programmation pluriannuelle de l'énergie pour la Guyane prévoit une évolution majeure du mode de traitement des déchets ménagers et assimilés pour la part non recyclable sous forme de valorisation énergétique en vue de produire de l'électricité. d'une nouvelle installation de stockage de déchets est en tout état de cause nécessaire, l'implantation d'une unité de valorisation énergétique des déchets est susceptible de rencontrer les mêmes difficultés juridiques. L'amendement n° 557 vise à la prise en compte des spécificités territoriales de la Guyane pour la mise en oeuvre de la loi Littoral, afin de permettre l'implantation d'installations de traitement des déchets tout en conservant le même niveau de protection du littoral. La Guyane est en effet confrontée à de nombreuses difficultés en matière de traitement des déchets. Du fait de la saturation prochaine de la décharge de Cayenne, il est urgent de lever les multiples contraintes législatives liées aux spécificités du territoire guyanais. Les contraintes liées aux risques aéroportuaires et à la loi Littoral empêchent toute création d'installations de traitement des déchets dans une zone accessible et à proximité des lieux de production des déchets. Si je suis favorable à l'amendement sur le fond, il est toutefois nécessaire d'apporter deux corrections mineures à sa rédaction d'une part, pour tenir compte du statut de la Guyane, qui n'est pas uniquement un département, et, d'autre part, pour déplacer la mesure dans la section spécifique à l'outre-mer des dispositions d'urbanisme de la loi Littoral.

Afin d'insuffler une dynamique au sein de l'État, des collectivités territoriales et des établissements hospitaliers pour tendre vers une consommation plus vertueuse des ressources disponibles, le présent amendement prévoit que les agents des trois fonctions publiques, ainsi que les élus locaux, puissent suivre une formation en matière d'économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets. La parole est à M.

Il précise les modalités sont lesquelles l'État assure la mission de suivi et d'observation des filières soumises à responsabilité élargie des producteurs ainsi que la communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets. Il renforce et complète le régime des sanctions pénales et administratives applicables aux acteurs des filières relevant de la responsabilité élargie des producteurs et à la lutte contre les gaspillages. Il vise également à renforcer l'efficacité de la police des déchets.

Il est grand temps d'en finir avec cette méthode antidémocratique qui consiste à légiférer toujours davantage par voie d'ordonnances et à faire passer la représentation nationale au second plan. Quel

l'indice de réparabilité était initialement annoncée pour 2020, il est donc aujourd'hui urgent de mettre en oeuvre cette mesure attendue par les consommateurs, qui souhaitent une information claire, nette et précise leur permettant de distinguer les produits les plus réparables.

d'outre-mer que pour celles de l'Hexagone. Les soutiens financiers versés par les éco-organismes, qui sont calculés en fonction des coûts observés en métropole, sont aujourd'hui très éloignés des coûts supportés par les collectivités d'outre-mer. Par exemple, alors qu'en moyenne les coûts réels supportés par les collectivités métropolitaines pour la collecte séparée et le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques sont couverts à hauteur de 50 % par les soutiens financiers des éco-organismes, ils ne le sont pour les collectivités d'outre-mer. L'obligation de mettre en place un barème de soutien financier majoré pour les collectivités d'outre-mer prévue par le présent projet de loi constitue donc une avancée majeure. Toutefois, la rédaction actuelle prévoit que l'application de ce barème spécifique ne sera obligatoire qu'au renouvellement de l'agrément des différents éco-organismes concernés, en 2023 pour les emballages ménagers, voire, au mieux, en 2021. Pourtant, le barème de soutien financier actuel est très insuffisant pour couvrir les coûts des collectivités d'outre-mer.

Jean-Louis Lagourgue. Dans les installations nucléaires de base, les INB, un zonage strict des déchets est établi. Il permet de distinguer deux types de zones : les zones « nucléaires » à production possible de déchets radioactifs

En effet, les opérations de démantèlement des installations nucléaires engendreront un volume important de déchets radioactifs, estimé à environ 2,3 millions de mètres cubes. Considérant les enjeux dans la perspective du démantèlement à venir, l'étude d'une méthode alternative au stockage qui permette de traiter ces déchets de manière fiable

faible activité, la perspective du démantèlement des installations nucléaires changeant les ordres de grandeur des volumes concernés. Différentes pistes, dont celle de recycler une partie de ces déchets, ont été étudiées dans le cadre du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs et sont actuellement évoquées dans le cadre du débat public préparant la future édition de ce plan.

indique clairement que « la consigne pour réemploi des emballages verre re-remplissables par rapport à l'utilisation d'emballages verre à usage unique présente toujours, dans le circuit des cafés, hôtels et restaurants, un gain environnemental qui se traduit par une baisse des émissions de gaz à effet de serre, des émissions de polluants dans l'air et dans l'eau,

Le scrutin est ouvert.

du territoire et du développement durable avait émis un avis défavorable sur ces amendements, mais qu'aucun scrutin public n'avait pour autant été organisé. Il me paraît nécessaire de pouvoir délibérer en toute responsabilité, publiquement, et avec vous, sur ces points essentiels.

ou les ampoules médicamenteuses emballées dans des plastiques opaques pour les protéger de la lumière et, par là même, assurer la sécurité sanitaire et médicale des patients.

! Vous dites que vous ne voulez pas détricoter le projet de loi. En fait, vous ne voulez pas le faire dans le cadre d'un débat démocratique à l'Assemblée nationale.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

il faut accompagner la volonté de nos concitoyens, qui souhaitent mieux consommer, ce qui passe évidemment par l'éducation dès le plus jeune âge et, surtout, par l'accès aux informations relatives aux caractéristiques environnementales des produits, ainsi qu'à leur durabilité.

tout en gardant en tête que l'économie était, il n'y a pas si longtemps, spontanément circulaire, et que la question du gaspillage ne se posait même pas. Ne le perdons pas de vue : si la loi est une chose, le marché en est une autre.

collectivement, du travail accompli. La création au sein de ce texte d'un titre spécifique pour donner un cadre juridique à l'État en vue de réduire drastiquement la production et la consommation de plastique est un bon exemple de notre travail transpartisan. Nous avons renforcé les droits du citoyen consommateur, valorisé le secteur du réemploi et l'économie sociale et solidaire, créé de nouvelles filières REP. Nous avons enfin défendu le service public des déchets,

remercier une nouvelle fois l'ensemble de l'hémicycle de la qualité de notre travail en faveur du nouveau paradigme circulaire dont notre système économique et notre planète ont tant besoin : cette nouvelle ère correspond mieux aux attentes des Français. Français. Enfin, en dépit des derniers épisodes que nous avons vécus, au terme de quatre journées d'intenses débats, il faut sortir de l'affichage et entrer dans le concret ; la balle est dans le camp du Gouvernement, mais nous voterons en

durable. Je dirai quelques mots, même si la plupart de mes collègues, et je les comprends, ont hâte de quitter cet hémicycle et de regagner leurs beaux départements respectifs.

suivie d'un débat, en application de l'article 50-1 de la Constitution, sur la politique migratoire de la France et de l'Europe, initialement prévue le mercredi 2 octobre à seize heures trente. Acte est donné de cette demande. En conséquence, le débat sur les conclusions du rapport d'information « Sécurité des ponts : éviter un drame » se tiendra le mercredi 2 octobre à partir de seize heures trente. Mes chers collègues, je constate que le Sénat a épuisé son ordre du jour pour la seconde session extraordinaire- s'il n'a pas épuisé les sénateurs et les sénatrices ! M. le président du Sénat prendra acte de la clôture de cette session lorsque nous aurons reçu le décret de M. le Président de la République portant clôture de la session extraordinaire du Parlement.